La séance est reprise. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif visant à sécuriser et réguler l’espace numérique est parvenue à l’adoption d’un texte commun. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la mise en place et au fonctionnement de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement

le niveau inédit de nos efforts en matière de solidarité internationale nous oblige, plus que jamais, à rendre compte de notre action en matière d’aide publique au développement et à l’évaluer. Après plusieurs années de baisse de notre aide publique au développement (APD), la France a engagé en 2017 un processus de refondation de sa politique de développement, afin de renforcer la crédibilité de notre action diplomatique, de répondre aux grands enjeux mondiaux et de maximiser l’impact de nos actions.

Avec près de 15,2 milliards d’euros en 2022, nous avons ainsi légèrement dépassé l’objectif intermédiaire, fixé par la loi du 4 août 2021, de 0,55 % du revenu national brut en 2022. tenu un engagement pris de longue date par le Président de la République. Les récentes annonces budgétaires ont toutefois une incidence sur la mission « Aide publique au développement », qui est mise à contribution comme toutes les politiques publiques.

Si les moyens que nous déployons sont inédits, ils ne permettent pas, à eux seuls, de répondre aux besoins et aux crises. Tel était le constat de départ du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial, qui a permis de mobiliser la communauté internationale face au défi du financement de la lutte contre la pauvreté et de la préservation de la planète. Nous continuons de porter cette ambition au sein des enceintes multilatérales et auprès de nos partenaires, grâce au pacte de Paris pour les peuples et la planète, aujourd’hui soutenu par cinquante quatre

lors d’une réunion du conseil présidentiel du développement, de dix objectifs prioritaires afin d’orienter notre action. Le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid) de juillet 2023 a ensuite permis de préciser les modalités de mise en œuvre de ces dix objectifs. Ces deux échéances majeures ont permis d’acter un changement de paradigme : la politique d’aide publique au développement s’est transformée en stratégie d’investissement solidaire. Ce choc de méthode doit permettre de rendre notre action plus efficace. La mise en œuvre de cette stratégie passe par un pilotage politique renforcé de nos actions. Celui ci n’est pas remis en cause par les récentes décisions budgétaires. Les priorités sont donc claires ; le cap est bien fixé. Je l’ai dit, l’efficacité de notre politique dépendra de l’évaluation des effets de nos actions. Si le Cicid a décidé que les ministres des affaires étrangères et de l’économie assurent l’évaluation de la mise en œuvre de nos priorités politiques dans le cadre d’une réunion annuelle, la loi de 2021 prévoit pour sa part la mise en place d’une commission indépendante d’évaluation de l’aide publique au développement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, n’ayez aucun doute quant à la volonté du Gouvernement de voir cette commission commencer rapidement ses travaux. Je tiens également à rappeler que, sur ce dossier, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a rempli ses obligations et assumé son rôle de chef de file de l’action extérieure. L’objectif L’objectif de la proposition de loi que vous examinez est simple : d’une part, débloquer la mise en œuvre de cette mesure importante de la loi de 2021 ; d’autre part, confirmer les missions de cette commission. Je me permets d’insister : il est bien question d’évaluer les projets et les programmes, et non pas simplement de contrôler l’usage des fonds. Dans cette perspective, nous acceptons volontiers que cette commission d’évaluation soit hébergée au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, et, comme nous l’avons confirmé à votre rapporteur, que le secrétariat administratif de la commission soit rattaché à la direction générale de la mondialisation,

des moyens humains et financiers supplémentaires seront affectés à cette commission, car sa tâche, d’ampleur – vous le concevez bien –, est à la mesure de l’effort inédit que je relevais en introduction de mon propos, de la richesse de nos coopérations et de la densité de nos échanges. Enfin, l’évaluation doit être envisagée comme un outil au service de l’amélioration de notre action, ainsi qu’au service de la France et de nos partenaires diplomatiques partout dans le monde. Les investissements réalisés aujourd’hui répondent à des besoins vitaux dans les pays bénéficiaires. Cependant, ils s’inscrivent aussi dans le temps long, car ils se concentrent sur des infrastructures stratégiques. Grâce à ces investissements, les populations sont mieux armées pour faire face aux conséquences du dérèglement climatique ; ainsi, l’accès à une source d’énergie décarbonée n’est pas réservé à quelques pays. Il est crucial que nos concitoyens prennent conscience que nos actions en faveur du climat, de la santé et de l’agriculture, partout dans le monde, contribuent également à leur avenir et à celui de leurs enfants.

La mise en place rapide de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement contribuera à l’efficacité de notre politique d’investissements solidaires. C’est pourquoi je vous invite à adopter ce texte. La parole

nécessaire, parce que l’aide publique au développement avait connu une progression considérable au cours des années précédentes. En particulier, les engagements financiers de l’Agence française de développement (AFD), principal opérateur de cette politique, étaient passés de 6 milliards d’euros en 2009 à 14 milliards d’euros en 2020. Une telle croissance a exigé de nombreux recrutements, mais aussi un élargissement de l’aide à un nombre considérable de pays. L’AFD a prospecté dans le monde entier pour placer ses prêts, souvent à des taux proches de ceux du marché, auprès de pays qui – il faut bien l’avouer – n’en avaient pas toujours un besoin évident.

De cette progression sans précédent des moyens et de cette expansion géographique permanente, il ne pouvait résulter qu’une demande accrue de contrôle et d’évaluation. est par essence difficile d’appréhender l’efficacité d’une politique de solidarité internationale. Ses projets sont, par définition, mis en œuvre dans d’autres pays que le nôtre, font souvent appel à des acteurs locaux et bénéficient à des populations dont notre connaissance est nécessairement limitée. À tort ou à raison, et malgré la qualité bien reconnue de nos opérateurs, ces projets soulèvent donc parfois des interrogations ou des doutes quant à leur efficacité, voire quant à leur bien fondé.

Il existe actuellement trois organismes d’évaluation interne en matière d’aide au développement, respectivement au sein du ministère de l’économie et des finances, du Quai d’Orsay et de l’AFD Concrètement, les évaluations pilotées par ces services sont réalisées par des cabinets de conseil sélectionnés par appels d’offres, sous la direction d’une équipe de responsables administratifs des ministères concernés ou de l’AFD.

Sénat. Toutes ces évaluations sont sans doute intéressantes et pertinentes. Cependant, un consensus s’est établi sur le fait qu’elles ne suffisaient pas à rendre compte de notre politique de solidarité internationale. D’abord, si les évaluations internes sont bien informées, elles aboutissent parfois à des conclusions stéréotypées et peu incisives, faute d’indépendance par rapport aux administrations ou aux opérateurs qui mettent en œuvre l’aide publique au développement. En outre, elles ont du mal à surmonter l’éclatement du pilotage de cette politique entre deux ministères et un établissement public. De plus, les évaluateurs externes ne disposent pas toujours des données ou des analyses nécessaires pour produire les évaluations les plus pertinentes.

Enfin, c’est la nature même des évaluations réalisées qui paraît insatisfaisante. Les instances d’évaluation actuelles concentrent souvent plus leur analyse sur les processus de gestion, l’organisation institutionnelle et les enjeux financiers ou budgétaires, que sur l’impact final et la pérennité des interventions françaises comme de l’influence de notre pays. C’est pour remédier à toutes ces limites que nous avons créé la commission d’évaluation indépendante, compétente de manière transversale pour l’ensemble des projets et des programmes de développement. Cette commission s’inspire de la commission indépendante pour l’impact de l’aide, ou (ICAI), mise en place au Royaume Uni, qui est composée de spécialistes du sujet, capables d’évaluer l’impact final des projets.

au millefeuille administratif. Dès lors, il fallait bien adosser la commission à une administration préexistante, apte à en assurer le secrétariat.

dont le Premier président, qui aurait logiquement présidé le nouvel organisme. Cette solution nous éloignait un peu du projet initial, qui consistait à créer un organisme, plus tourné

Cet adossement administratif au ministère chargé des affaires étrangères paraît finalement le plus simple à mettre en œuvre, donc le plus propre à permettre le lancement rapide des travaux de cette commission, que nous attendons tous depuis plus de deux ans. Je rappelle que la loi dispose toujours que les experts de la commission sont indépendants et qu’ils déposent une déclaration d’intérêt. En outre, n’oublions pas la présence

nous avons déjà commencé nos échanges avec l’administration sur ce sujet. De même, nous espérons qu’une personnalité indépendante, d’une expertise reconnue en matière d’aide publique au développement, sera élue à la tête de la commission ; nous estimons qu’il doit s’agir d’un emploi à temps plein.

la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui nous permet, enfin, de sortir de l’ornière. Ce texte reste en outre très proche de la loi de 2021 que nous avions votée, je le rappelle, à l’unanimité. C’est pourquoi la commission l’a adopté sans modification. Nous espérons ainsi mettre le point final à un feuilleton qui n’aura que trop duré, pour doter enfin notre politique de solidarité internationale d’une instance d’évaluation digne de ce nom, dans laquelle le Parlement jouera, à l’évidence, un rôle très important. La parole

Il a permis de porter les crédits alloués à l’aide publique au développement à 0,55 % du revenu national brut en 2022, conformément à l’engagement du Président de la République, avec l’objectif d’atteindre 0,7 % en 2025.

Autre exemple, un manège a été installé devant la maison de la Russie à Bangui. J’y ai vu une belle illustration du fait que le Kremlin cherche à faire tourner les Africains en rond ! La mission de notre aide publique au développement est plutôt de bâtir un monde à la fois plus juste et plus durable. Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance : les équipes de l’AFD sont engagées dans plus de 4 000 projets dans 150 pays, contribuant ainsi à l’engagement de la France en faveur du développement durable et du respect de l’accord de Paris. Tel est l’objectif qui doit étayer notre politique de développement. Lors de l’examen des crédits de la mission « Aide publique au développement », plusieurs de nos collègues avaient insisté sur la nécessité de se doter de mécanismes susceptibles d’améliorer le contrôle et le suivi des aides accordées par notre pays. C’est non seulement un enjeu d’efficacité, mais également une nécessité au regard du contrôle démocratique que doivent exercer les assemblées parlementaires en général et le Sénat en particulier. La France a mis en œuvre de nombreux projets au travers de la politique de l’AFD. Souvent, j’ai pu juger sur place de leur réussite. Ainsi, j’ai participé l’an dernier, à Antananarivo, à la cérémonie d’inauguration du parcours touristique de la Haute Ville, en présence du ministre malgache de l’aménagement du territoire, du maire de la capitale et de notre ambassadeur. Cette véritable réussite urbanistique avait pour but de désenclaver et d’assainir des quartiers prioritaires. Lors de la visite, revêtu de mon écharpe tricolore, j’ai observé les sourires des habitants qui profitaient de points d’eau et de lavoirs flambant neufs. Quelle fierté d’avoir été accompagné par une partie des habitants durant cette déambulation et de les avoir entendus crier : « Vive la France ! » L’aide publique au développement constitue un outil efficace et essentiel au service de la stratégie d’influence de notre pays. Nous devons assumer cette ambition sans naïveté, comme de nombreux autres pays le font. La loi de programmation du 4 août 2021 avait mis en place une commission d’évaluation des politiques d’aide publique au développement, ce qui répondait à une demande que le Parlement, particulièrement le Sénat, formulait depuis de nombreuses années. Deux ans après la promulgation de cette loi, la commission d’évaluation de l’aide publique au développement n’est toujours pas constituée, les modalités de son rattachement à la Cour des comptes et de la désignation de son président étant encore en suspens.

La nécessité de bien évaluer l’aide paraît plus prégnante que jamais, compte tenu de l’augmentation des moyens de cette politique, passés de 9,5 milliards d’euros à près de 15 milliards d’euros entre 2016 et 2023. Dans son rapport au Premier ministre d’août 2018 sur la modernisation de la politique partenariale de développement, M. Hervé Berville, rapporteur de la loi du 4 août 2021 à l’Assemblée nationale, plaidait pour que l’évaluation devienne un axe central de notre politique de partenariats et de solidarité internationale. Nous souscrivons à cette analyse. Un cadre d’évaluation adéquat et une diffusion de la pensée évaluative sont de nature à améliorer l’efficacité de l’action publique et à renforcer les partenariats avec les pays concernés. Ils offrent aussi l’occasion d’un dialogue approfondi sur les objectifs stratégiques et la définition d’attentes communes, ainsi que la recherche d’un consensus. Dans cette optique, l’indépendance de la commission est absolument capitale.

L’article 2 du décret n° 2022 787 du 6 mai 2022 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d’évaluation de l’APD précise la composition du collège d’experts. Le décret précise également que la commission élit son président à l’unanimité parmi ses membres, ce qui, en pratique, aurait conduit à l’élection du Premier président de la Cour des comptes. cette composition ne répond pas à la volonté du législateur de créer un instrument nouveau chargé d’évaluer les projets de développement et non de contrôler leur régularité financière. Clairement, les résultats de l’APD ne peuvent se mesurer seulement,

Nous aussi, parlementaires, devons mouiller l’écharpe tricolore en inaugurant les projets financés par l’AFD ! Les investissements de la France auprès de nos partenaires se mesurent également à l’aune de leur effet sur les populations, ainsi que du rayonnement et de l’influence de notre pays. de loi que nous examinons permet de rattacher la commission d’évaluation au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, pour ce qui a trait à son fonctionnement. Le texte précise aussi les missions assignées à cette commission.

Ce sont la fraternité et la sororité qui réconcilient le désir de liberté et l’exigence d’égalité. Ce sont la fraternité et la sororité qui permettent de créer du lien malgré nos diversités d’origine, de croyance et de culture. Surtout, ce sont la fraternité et la sororité qui permettent la solidarité et le partage entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n’ont pas assez. Alors qu’aujourd’hui les pays de l’OCDE affichent un revenu par habitant cinquante deux fois supérieur à celui des pays à faible revenu, alors que la moitié de la population mondiale n’a pas accès aux services de santé essentiels, alors que les impacts du dérèglement climatique sont de plus en plus visibles et destructeurs et qu’il existe un problème d’accès à l’eau pour un grand nombre de populations, la France doit continuer à faire rayonner ces valeurs de fraternité et de sororité, piliers de notre promesse républicaine, au moyen de l’aide publique au développement. Cependant, elle doit le faire avec éthique, équité et transparence.

solidaire et durable, en se fixant des objectifs à l’horizon de 2030. À mi parcours de cette échéance, deux ans après l’adoption par le Parlement de la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, il est nécessaire de dresser un bilan de rappeler le contexte, ainsi que la philosophie dans laquelle doit s’inscrire notre action en la matière, afin de voir comment nous pouvons gagner en efficience et en transparence. Tout d’abord, au regard de l’accentuation des inégalités, je tiens à saluer l’engagement pris par notre pays d’allouer 0,55 % du revenu national brut à l’APD. Cet engagement, pris devant les instances internationales, symbolisait la volonté de la France de contribuer de manière significative à l’effort global de développement. Malheureusement, aujourd’hui, cet engagement n’est pas tenu.

Cette incohérence entre nos engagements et les annonces du Gouvernement écorne l’image de notre pays, d’autant que nous avons organisé, pas plus tard qu’en juin dernier, un sommet ambitieux pour un nouveau pacte financier et un plan de bataille mondial de réduction de la pauvreté et de lutte contre le changement climatique. Il est urgent de respecter notre promesse, car un manquement apparaîtrait comme un renoncement à notre responsabilité vis à vis du monde et, plus particulièrement, des pays les plus vulnérables. alors que la France a connu de nombreuses difficultés sur la scène internationale, notamment en Afrique, un tel renoncement serait perçu comme un énième signe de faiblesse envoyé à ceux qui aimeraient voir notre pays s’affaisser au niveau d’une puissance moyenne du point de vue géopolitique.

En Afrique, il est nécessaire de nous projeter vers l’avenir, de reconnaître et d’assumer notre histoire coloniale. L’APD est l’un des moyens grâce auxquels nous pouvons contribuer à réparer les séquelles laissées par des siècles de domination. Il s’agit non pas de charité, mais de justice et de reconnaissance des interdépendances qui nous lient à ces pays. En privilégiant des projets qui soutiennent l’autonomie et le développement durable, en écartant toute forme de néocolonialisme économique, nous poserons les bases d’un nouveau partenariat qui marquera le retour de la France. que la nécessité des financements s’est accrue, une attention particulière doit être accordée aux pays les moins avancés, avec une préférence pour les dons plutôt que les prêts. En effet, ces derniers, bien que parfois nécessaires, accroissent l’endettement des pays bénéficiaires, les enfonçant dans un cycle de dépendance et de vulnérabilité financière. Cette situation est préoccupante, dans un contexte où de nombreux pays en développement luttent déjà contre des défis économiques majeurs, exacerbés par le réchauffement climatique et les crises. (Cese), je recommande que la France promeuve l’adoption de nouvelles sources de financement innovantes, ainsi que l’augmentation des recettes de taxes existantes consacrées au développement des pays les moins avancés, comme la taxe sur les transactions financières ou la taxe de solidarité sur les billets d’avion.

dans un souci de plus grande cohérence, on nous propose de placer cette commission sous l’autorité du ministre des affaires étrangères. Les arguments en ce sens se tiennent et nous pouvons entendre cette logique, mais cela ne saurait se faire au détriment des exigences de transparence, d’équité et d’indépendance.

dans le consensus parlementaire cristallisé dans la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

le Président de la République a décidé, arbitrairement, lors du conseil présidentiel du développement qu’il a réuni en mai 2023, de modifier toutes les orientations de la loi de 2021. Le comité interministériel de la coopération internationale et du développement a pris acte des orientations du Président et a notamment décidé, en juillet dernier, de modifier les objectifs de l’APD, alors même que ces derniers avaient été inscrits dans la loi adoptée deux ans plus tôt.

Une telle baisse de l’APD est incompatible avec les engagements de la France et avec son action diplomatique. Gardons nous de faire perdre à la France sa crédibilité sur la scène internationale Pourtant, des solutions existent, comme la taxe sur les transactions financières. Pourquoi celle ci reste t elle plafonnée à 528 millions d’euros, alors même que son objectif initial était de participer à la solidarité internationale ?

augmentons massivement le volume de notre fonds de solidarité pour le développement en rehaussant le taux de la taxe sur les transactions financières de 0,3 % à 0,7 % et en élargissant son assiette, afin que plus d’entreprises y soient assujetties.

on parle de 15 milliards d’euros par an, d’un budget qui a progressé d’un tiers depuis 2017 et d’une situation internationale extrêmement préoccupante dans de nombreuses régions du monde. Dans le même temps, cette politique publique, à tort ou à raison, tend à devenir un outil supplémentaire au service de notre diplomatie, dans un contexte – il faut bien le reconnaître – de déclin de notre rayonnement et de notre influence. Analyser l’impact de nos financements ici ou là dans le monde n’est pas un luxe. Face aux « narratifs » de nombreux états hostiles à la France et à l’Occident, le soutien que nous apportons un peu partout mérite d’être connu et reconnu. Une démarche d’évaluation ne peut être qu’utile et porteuse de progrès. En outre, on l’a vu récemment, les crédits affectés à l’aide publique au développement sont toujours, quelle que soit l’ambition de départ, une cible facile pour les coupes budgétaires. Le décret d’annulation de crédits du mois dernier ôte 742 millions d’euros à l’APD, premier poste raboté en pourcentage. Or, beaucoup plus que par le passé, cette politique publique engage désormais la stabilité, la sécurité et la paix.

La mise en place de cette commission devait permettre, dans l’esprit du législateur, de conduire des évaluations portant sur l’efficience, l’efficacité et l’impact des stratégies, des projets et des programmes d’aide publique au développement financés ou cofinancés par la France. Le ministre des affaires étrangères serait donc juge et partie ; ce n’est pas judicieux, car il faut garantir l’indépendance de la commission. Il était pourtant si facile de rattacher cette commission au Parlement,

Autre regret pour le groupe du RDSE : aucun échange formel n’est prévu entre les collectivités territoriales et la commission d’évaluation. C’est dommage, car la coopération décentralisée a des choses à nous apprendre. C’est aussi le sens d’un amendement de notre collègue Rachid Temal. état de cause, ce texte s’inscrit dans une nécessité temporelle et il faut avancer. Le RDSE fera le choix du pragmatisme : ses membres voteront pour ce texte afin de permettre, après deux longues années d’attente, l’institution effective de cette commission.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la France figure parmi les plus grands contributeurs mondiaux à l’aide publique au développement. Plus de 15 milliards d’euros y ont été consacrés par C’est bien sûr un motif de satisfaction pour la France, mais cela nous donne également une grande responsabilité quant à la manière dont cette aide est employée. En 2021, nous avons adopté une loi destinée à encadrer l’aide publique au développement. À cette occasion, nous nous sommes fixé un objectif quant au montant que notre pays devait lui La France devra lui allouer en 2025 0,7 % de son revenu national brut ; il s’agit du seuil préconisé par les Nations unies. La France progresse vers cet objectif, malgré les difficultés budgétaires auxquelles elle est confrontée. En temps de crise, la tentation est grande pour les États donateurs de faire l’impasse sur l’aide au développement, mais c’est précisément dans de telles périodes que cette aide est encore plus nécessaire aux populations qui en bénéficient. Notre groupe soutient une conception de l’aide au développement tournée vers les partenariats et l’investissement. Nous approuvons la volonté exprimée par le chef de l’État de conduire des projets en traitant directement avec les sociétés civiles. Enfin, nous tenons à ce que l’aide accordée par la France, issue de l’argent du contribuable, soit étroitement contrôlée. Nous devons nous assurer qu’elle ne bénéficie en aucune manière à nos adversaires et nous devons garantir l’efficacité de notre aide, afin que chaque euro compte. 4 août 2021 prévoyait de renforcer ce contrôle par la création d’une commission. Il est prévu que cette commission d’évaluation transmette des rapports annuels au Parlement afin de mieux éclairer ce dernier sur les conséquences de l’aide publique dont il vote chaque année les crédits. trois ans après l’adoption de cette loi, ladite commission n’a pas encore pu se réunir. Sa mission n’a pas été définie avec suffisamment de précision. La publication du décret du 6 mai 2022 a laissé entrevoir une restriction de sa mission d’évaluation de l’aide publique. La commission s’apparentait de plus en plus à une commission de contrôle budgétaire. Sa présidence aurait ainsi été confiée, dans les faits, au Premier président de la Cour des comptes. Or l’évaluation de la pertinence de l’aide publique de notre pays ne peut valablement se faire au travers du seul prisme budgétaire. L’examen financier est bien entendu nécessaire, mais il est insuffisant. Nos collègues députés nous proposent aujourd’hui de préciser la mission de la commission d’évaluation. Celle ci ne devra pas se contenter de rendre des avis budgétaires, mais aussi apprécier la conformité des projets financés aux besoins identifiés des populations, ainsi qu’aux intérêts de la France, l’aide publique au développement accordée par notre pays doit servir nos intérêts – il serait bien naïf d’agir différemment. Les auteurs du texte proposent de rattacher la commission non à la Cour des comptes, mais au ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Ce rattachement nous paraît plus cohérent avec les objectifs de la commission. Plusieurs dispositions du texte garantissent en outre l’indépendance des experts de la commission d’évaluation, qui seront tenus de remplir des déclarations d’intérêts afin de prévenir tout conflit en la matière. la commission des affaires étrangères, le rapporteur Christian Cambon a proposé une adoption conforme du texte. Nous ne pensons pas qu’il soit opportun d’ouvrir d’autres débats relatifs à l’aide publique au développement. Nous sommes également persuadés qu’il est nécessaire de régler la question de cette commission d’évaluation au plus vite, afin de lui permettre de se réunir et de commencer à travailler. Aussi n’avons nous pas déposé d’amendement. Le groupe Les Indépendants – République et Territoires soutiendra l’adoption de cette proposition

au cœur de l’été 2021, le Parlement votait, à une rare unanimité des groupes politiques, la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Mes collègues l’ont rappelé, ce texte a rénové en profondeur le cadre de la politique française d’aide publique au développement, mais également sa philosophie.

définissait les priorités sectorielles et géographiques, renforçait les partenariats avec dix huit pays africains et Haïti et révisait le pilotage de l’aide au développement.

Première carence, qui était pourtant une mesure emblématique de la loi de 2021 : les conseils locaux de développement, institués au sein des ambassades pour produire des stratégies au plus près des réalités,

Dans d’autres postes diplomatiques, les conseillers des Français de l’étranger, qui doivent pourtant être associés à ces conseils, n’ont simplement pas été invités. En tant que sénateur représentant les Français de l’étranger, mais surtout en tant que conseiller des Français de l’étranger pour la Côte d’Ivoire et le Liberia, je ne peux que regretter ces oublis fâcheux. effet les conseillers des Français de l’étranger qui connaissent le mieux les écosystèmes, les populations locales, leurs spécificités et leurs besoins ; leur expertise est un atout précieux, dont il faut se servir. On peut regretter qu’aucun texte réglementaire n’ait été publié pour organiser le fonctionnement de ces conseils locaux. Deuxième carence, et non des moindres

Il s’agit de mener de façon indépendante une évaluation concrète et non uniquement financière – ce serait trop réducteur – de l’efficience, de l’efficacité et de l’impact des projets et des programmes d’aide publique au développement auxquels la France participe. Il faut impérativement passer d’une évaluation comptable à une démarche fondée sur la performance, sur le pilotage par les résultats, en se demandant par exemple combien de kilomètres de route ont été construits, combien de malades du paludisme ont été soignés, combien de classes ont elles été ouvertes, ou combien de filles et de femmes ont pu accéder à des protections hygiéniques. Voilà ce qui importe, voilà ce que nous devons mesurer Cette commission n’est donc en rien un énième comité Théodule, symptôme d’une pathologie française, symbole de l’impuissance du politique, mais un outil pertinent de pilotage et de contrôle d’une politique publique dont le budget, qui avoisine déjà 15 milliards d’euros, est appelé à croître au cours des prochaines années. Sa mise en place est donc urgente et indispensable à la réalisation de nos ambitions. La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à résorber les quelques blocages qui ont retardé sa création. L’inscription dans

Son placement auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, prévu par le texte, permet d’éviter ce glissement comptable. Le texte précise également les missions assignées à la commission. Elle évalue les projets et programmes d’aide publique au développement, depuis leur conception jusqu’à leur mise en œuvre. Les résultats sont évalués du point de vue financier, mais aussi au regard des orientations de la France en matière de politique extérieure et de coopération et des intérêts de la France à l’étranger. Ces clarifications me semblent de bon aloi, car elles placent l’aide publique au développement dans un cadre de réflexion stratégique plus global. Cela étant, je souhaite porter à l’attention des futurs membres de la commission d’évaluation deux points qui me semblent d’importance. Le premier point concerne le détournement des flux d’aide au développement. Ce phénomène, que beaucoup préfèrent minimiser, voire ignorer, existe bel et bien, même s’il est difficile à évaluer. La Banque mondiale s’y est essayée en 2020. En ce qui concerne les vingt deux pays les plus dépendants de son aide, elle estime à au moins 5 % la part des flux détournés vers des paradis fiscaux. Ces fuites dans l’organisation de l’aide viennent renforcer des régimes corrompus ; la captation indue des richesses appauvrit encore davantage les populations et entrave le développement.

Nous connaissons tous les débats sur la tutelle de l’AFD, je n’y reviendrai pas. Dans son discours de clôture des États généraux de la diplomatie, il y a un an, le président Macron Macron rappelait que l’AFD est l’outil essentiel de la France en matière de gestion des fonds publics destinés à l’aide publique au développement. Il avait néanmoins souligné la nécessité, pour l’Agence, de travailler en synergie et en bonne intelligence avec le ministère des affaires étrangères et de l’Europe de déployer des partenariats stratégiques, venant ainsi appuyer les recommandations que la Cour des comptes avait formulées dans sa note d’analyse de février 2020. de février 2020. Cette commission d’évaluation me semble être en droite ligne avec cet objectif. Elle encouragera en effet les relations entre l’AFD et le MEAE. Son rattachement au ministère s’impose logiquement. La commission d’évaluation doit incarner tout ce qui précède. Il faut conclure, cher collègue. Elle saura porter avec beaucoup de sérieux l’exigence nécessaire à ce travail. Nos quatre collègues députés et sénateurs veilleront au respect de l’esprit qui anime nos débats. Pour l’ensemble des raisons que je viens d’évoquer, je souscris entièrement aux dispositions de cette proposition de loi, que je voterai sans réserve. Merci

Le texte précise que cette commission est chargée de l’élaboration d’un « cadre d’évaluation permettant de mesurer l’efficacité et l’impact de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales En 2022, la France a consacré à 15,2 milliards d’euros à l’aide publique au développement, faisant de notre pays le quatrième bailleur mondial en matière d’aide

La création d’une commission d’évaluation spécifique répond parfaitement à cette demande, formulée par souci d’efficacité. En effet, la commission aura pour mission d’assurer la traçabilité et l’efficacité de notre aide publique au développement. Je précise, comme certains d’entre vous l’ont fait avant moi, que cette évaluation ne se fera pas uniquement à l’aune de critères financiers. Très simplement, il ne s’agit pas de dire si l’argent public est bien dépensé ou non. Le travail de la commission prendra en compte un certain nombre de paramètres, comme le respect des dix objectifs fixés par le Conseil présidentiel du développement, qui s’est tenu l’année dernière. Ce travail d’évaluation sera minutieux. Il s’agira de scruter l’avancée des projets d’aide publique au développement et de se poser des questions on ne peut plus concrètes. Les droits humains sont ils bien protégés au Brésil ? L’accès à la santé a t il été dûment garanti au Liban ? Combien de femmes auront elles bénéficié du plan de lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales

L’Agence française de développement est devenue une véritable plateforme pour le développement. Je tiens à cette occasion à saluer le travail formidable qu’elle réalise. Les femmes et les hommes qui travaillent à l’AFD contribuent à traduire en actions notre politique de développement dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’environnement, et dans bien d’autres encore. La commission d’évaluation de l’aide publique au développement rendra justice à l’immense travail qui est mené. Elle permettra également aux grands acteurs du développement de renforcer leurs exigences, ce qui affinera davantage la qualité de leur activité.

Je l’ai dit à cette tribune, lors de nos débats sur le projet de loi de finances pour 2024 : accompagner les pays les plus fragiles, c’est assurer notre propre sécurité. Les ressources que nous allouons à notre politique de solidarité internationale ont un double effet. Elles servent à la fois un objectif de développement et un objectif de diplomatie. L’aide publique au développement permet le développement et l’entretien de relations bilatérales saines avec de nombreux pays. Quant à la qualité de ces relations, elle renforce la stabilité mondiale. Malgré son importance capitale, notre politique de développement est mal connue du grand public. La commission d’évaluation garantira plus de visibilité à notre action. Cette commission est, somme toute, absolument nécessaire à la mise en œuvre et à la bonne compréhension de l’aide publique au développement. Cependant, cette commission n’a toujours pas été instituée, trois ans après la promulgation de la loi de 2021, en raison de la confusion créée par le décret du 6 mai 2022 relatif à ses modalités de fonctionnement. Comme vous Comme vous le savez, ce décret prévoit que sur les dix postes du collège d’experts indépendants, deux doivent être réservés à des magistrats de la Cour des comptes en activité, dont son Premier président. Sachant que ce même décret prévoit que le président de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement est élu par et parmi ses membres, il devenait presque naturel que le Premier président de la Cour des comptes devienne le président de la commission d’évaluation. je suis d’accord avec la proposition de loi sur le point suivant : ce décret pousse la commission d’évaluation sur un chemin qui n’a pas été tracé par le législateur, lequel avait certes confié le rattachement et le secrétariat de cette instance à la Cour des comptes, mais n’avait en aucun cas prévu

vise également à mettre fin aux blocages et à dissiper définitivement toute confusion, en rattachant la commission au ministère des affaires étrangères. Pilote principal de notre politique nationale d’aide publique au développement, le ministère des affaires étrangères ne sera toutefois que le ministère de rattachement de la commission Il n’exercera en aucun cas une tutelle sur celle ci. Bien au contraire, le ministère garantira l’indépendance de ses travaux. De plus, il gérera l’accueil et le secrétariat de la commission et veillera qu’aucun de ses membres ne soit en situation de conflit d’intérêts. Parce que cette commission d’évaluation est nécessaire à la conduite de notre politique d’aide au développement et qu’il est plus que temps qu’elle soit instituée, le groupe RDPI votera en majorité pour ce texte.

pour laquelle, cher collègue, nous avions distingué deux collèges, un collège d’experts et un collège de parlementaires : le collège d’experts était chargé d’expertiser les dossiers et de réaliser ce travail

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

au regard des ambitions et des objectifs prévus par la loi et elle en examine les résultats pour apprécier leur efficacité, tant sur le plan financier que vis à vis des priorités de la politique extérieure

des fonds. Monsieur le sénateur, vous avez participé, en tant que parlementaire, à la revue de l’aide publique au développement de l’OCDE. Vous savez donc que l’analyse de la pertinence est l’un des six grands critères

en raison des pouvoirs de sanction importants dont ils sont dotés et qui confèrent une importance particulière à leur déclaration d’intérêts. Il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, de tordre le cou au droit de la fonction publique.

Il est bien évidemment hors de question de se priver de l’avis des collectivités territoriales, comme cela a été souligné dans de nombreuses interventions. Pour autant, il ne me semble pas nécessaire de les mentionner dans la loi, car il faut au contraire, pour renforcer le travail de la commission

avec les différents volets des investissements solidaires et durables. Par ailleurs, les membres de cette commission sont désignés pour leur expertise et leur diversité. Outre les échanges conduits dans le cadre des travaux de la commission,

Par ailleurs, monsieur le sénateur, je vous rappelle, mais j’imagine que vous le savez, que deux instances de concertation avec les élus locaux et la société civile existent déjà : la Commission nationale de la coopération décentralisée et le Conseil national pour le développement et la solidarité internationale,

Nous verrons bien dans quelque temps ce que fera cette commission d’évaluation.

parole ?… Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi relative à la mise en place et au fonctionnement de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement instituée par la loi n° 2021 1031 du 4 août 2021. Je rappelle

professionnel français. Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux de pouvoir de nouveau réaffirmer ma volonté de frapper toujours plus fort les délinquants au portefeuille. La proposition de loi que nous examinons ce soir vise à renforcer nos capacités de saisies et de confiscations. Son objectif est clair : nul ne doit tirer profit de son crime. Je la soutiens donc avec force. Nous avons déjà renforcé notre arsenal avec la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, dite loi Warsmann. Avec cette loi, l’approche judiciaire a été rénovée. Les enquêtes ont connu une nouvelle dynamique. Les investigations ont dépassé le simple recueil de preuves de la commission d’une infraction ; elles sont devenues patrimoniales. Forte de ces investigations portant sur la composition du patrimoine des délinquants, notre action judiciaire a été renforcée. D’une part, les possibilités de saisies, au stade de l’enquête, ont été étendues à tous les biens « confiscables » afin que les juridictions de jugements puissent confisquer confisquer l’ensemble des avoirs criminels. D’autre part, l’État s’est doté, pour la première fois, d’un dispositif permettant de gérer les biens saisis et confisqués. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) a ainsi été créée. Cette agence est devenue le bras armé de l’État pour aller chercher réparation auprès des délinquants en les tapant directement au portefeuille. Ce bras armé, intégré à un nouvel arsenal, s’est révélé d’une efficacité redoutable. Les chiffres parlent d’eux mêmes.

Vous le savez, l’augmentation des saisies et des confiscations constitue un axe fort de ma politique pénale. J’ai demandé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République de conduire une politique pénale volontariste en favorisant la saisie et la confiscation des avoirs criminels. La mobilisation de mon ministère n’a jamais fléchi La confiscation des fonds, des comptes bancaires, des meubles et des biens immeubles des auteurs d’infractions a atteint des chiffres records. Chaque année, les policiers, les gendarmes, les douaniers, les procureurs de la République, les juges d’instruction et les juges des libertés et de la détention font preuve d’un engagement sans faille. Ils s’emparent plus fortement de cet outil précieux de lutte contre le crime. La confiscation du patrimoine des criminels est, en effet, un levier incontestable de la répression. Là encore, les chiffres relatifs aux confiscations sont éloquents. En 2020, le montant des confiscations prononcées par les juridictions pénales s’élevait à 86 millions d’euros. 2023, il atteignait 175,5 millions d’euros, soit une hausse de 105 % ! Pour intensifier cette politique pénale hautement stratégique, j’ai renforcé les capacités d’action de l’Agrasc. Désormais, l’Agence rayonne sur l’ensemble du territoire national, au plus proche des juridictions. Huit antennes régionales ont ainsi été créées : à Marseille, à Lyon, à Lille, à Rennes, à Bordeaux, à Nancy, à Fort de France et à Paris. L’efficacité de l’Agence le soutien qu’elle apporte aux juridictions ont ainsi été redoublés. Au plus près des enquêteurs et des magistrats, l’Agrasc leur dispense des conseils et les oriente. Les scellés sont mieux gérés et l’exécution des décisions de confiscation a gagné en efficacité. Surtout, nous avons considérablement renforcé les moyens humains de l’Agrasc. Vous le savez, ma politique au ministère de la justice est constante : si on veut des résultats, il faut y mettre les moyens ; et quand on a mis des moyens, il nous faut des résultats

par deux. Si la confiscation des avoirs criminels est l’une des armes de la répression, elle est également un levier efficace d’indemnisation et de réparation. Je veux ainsi souligner que désormais les biens immobiliers confisqués peuvent connaître une réaffectation sociale pour que puissent être développés des programmes d’intérêt public. Grâce à la loi du 8 avril 2021 rapportée au Sénat par votre collègue Alain Marc, des associations, des fondations ou des foncières solidaires, peuvent se voir attribuer des immeubles confisqués aux délinquants par nos juridictions pénales. Il y a un an, à Coudekerque Branche, j’ai remis les clés du premier immeuble saisi par la justice à l’association Habitat et Humanisme. Permettez moi de vous dire que, à mon sens, cette pratique incarne l’idée même de justice. Ce dispositif a été pensé dans une logique réparatrice, au service des victimes et des plus démunis. C’est par ce type d’actions fermes, efficaces, mais surtout justes, que nous retisserons le lien de confiance entre l’institution judiciaire et nos concitoyens. basculé dans une autre dimension, inspirée par les dispositions italiennes antimafia, qui nous permet de nous inscrire au plus proche des besoins des communes, au bénéfice direct de nos concitoyens. Trois immeubles ont ainsi été affectés socialement en 2022 : une villa confisquée par le tribunal correctionnel de Pointe à Pitre a été remise à une association chargée de prévenir la récidive en matière de violences conjugales ; l’immeuble confisqué par le tribunal correctionnel de Dunkerque, que j’évoquais précédemment, a été remis à une association pour y réaliser des logements sociaux ; un logement, confisqué par le tribunal correctionnel de Montpellier, a été réaffecté pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Enfin, un autre progrès permettant la restitution des biens mal acquis aux populations spoliées a été consacré par la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Désormais, le produit des biens confisqués dans le cadre des affaires dites de « biens mal acquis » par des dirigeants étrangers peut être affecté au financement de l’action de coopération et de développement, au profit des populations des pays concernés. Nous partageons tous le même constat : l’objectif des délinquants et des criminels ne repose pas sur des valeurs humanistes ; il est d’engranger du profit. Nous avons mis en place un cercle vertueux et les avancées sont incontestables, mais il nous faut encore aller plus loin et frapper plus vite, frapper plus fort le patrimoine des criminels et des délinquants. Car après une décennie de progrès, certaines lacunes ont été identifiées, qu’il convient de combler. Plusieurs recommandations du rapport de MM. Warsmann et Saint Martin de 2019 ont d’ores et déjà été mises en œuvre. Mais pour que le crime ne profite plus, il nous faut encore renforcer notre législation afin de consolider les actions judiciaires. Tel est l’objet de cette proposition de loi : il nous faut combler certaines failles, il nous faut parfaire un édifice, même s’il repose déjà sur des fondements solides. Il nous faut pouvoir saisir plus et confisquer mieux les produits des crimes, les profits générés par les délinquants. Je sais que cet objectif nous rassemble. les dispositions de la proposition de loi qui tendent à faciliter notamment les ventes avant jugement sont les bienvenues. Je veux d’ailleurs saluer les travaux de la commission, qui ont permis de préciser certaines dispositions et d’améliorer l’efficacité de l’arsenal proposé. L’article 1 prévoit d’accélérer la vente des biens saisis avant jugement en allégeant les modalités des voies de recours. La commission des lois et votre rapporteure, dont je veux ici saluer le travail, a étendu cette procédure simplifiée de recours à l’ensemble des saisies, ainsi qu’aux décisions de non restitution des biens. Elle a prévu, en outre, que la vente avant jugement des biens saisis pourra intervenir plus largement, notamment lorsqu’il s’agit de biens dont la valeur se déprécie rapidement ou qui engendrent des frais d’entretien trop importants. L’affectation sociale des biens immobiliers saisis a été étendue au profit notamment des services judiciaires et des services chargés de missions de police judiciaire. La procédure de convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) a été enrichie. La possibilité de contraindre les personnes morales à se dessaisir des biens saisis au profit de l’État les juridictions de jugement n’auront plus l’obligation de motiver la peine de confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction. La proposition de loi a été enrichie à l’issue notamment des travaux de la commission des lois de votre assemblée. Elle permettra de frapper mieux et plus vite les délinquants au portefeuille. L’article 2 a un objectif clair : améliorer l’indemnisation des victimes. Pour cela, les parties civiles pourront désormais obtenir le paiement de leurs dommages et intérêts non seulement sur les biens confisqués définitivement, mais également sur les biens dévolus à l’État et ceux ayant fait l’objet d’une décision de non restitution. Votre commission des lois a également prévu de permettre aux officiers de police judiciaire de procéder à une saisie élargie des patrimoines. Le régime prévu apporte à notre dispositif de saisie indispensable, qui visera également les sommes versées sur les comptes de paiement des néobanques. L’article 3 vise à renforcer l’efficacité des saisies en ne permettant plus que des proches du délinquant ou du criminel continuent de profiter des biens qui auraient été saisis par la justice. d’élargir le mécanisme de restitution des biens mal acquis, notamment aux sommes saisies et confisquées sur les comptes bancaires. Un cap a été franchi ces dernières années, les résultats des saisies et des confiscations sont inédits. La proposition de loi permettra messieurs les sénateurs, l’engagement du Gouvernement, et du ministère de la justice en particulier, pour lutter contre la délinquance et la criminalité est total. Il est temps ce soir d’aller plus loin pour que le crime ne paie pas, pour que le crime ne paie plus

et une proposition de loi avait été votée, mettant en place l’architecture générale de l’appréhension du patrimoine des délinquants. En 2019, le Premier ministre de l’époque avait confié à MM. Warsmann et Saint Martin

nous n’avons pas beaucoup d’influence sur cet aspect là des choses, il est extrêmement important que le système numérique permette le suivi des avoirs, de la saisie jusqu’à la confiscation.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le crime ne paie pas, ou en tout cas ne devrait pas payer. Le constat est simple d’ailleurs délinquance en col blanc, financière, liée au narcotrafic ou autre –, détestent être frappés au portefeuille. « Pour être véritablement dissuasive, toute sanction pénale doit pouvoir s’accompagner de la privation des délinquants des profits qu’ils ont pu tirer de l’infraction.

La confiscation est une peine complémentaire de plein droit pour les infractions punies d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse, et peut porter sur l’ensemble des biens ayant un lien avec un crime ou un délit, qu’ils aient servi à commettre l’infraction ou qu’ils en soient le produit direct ou indirect.

la rapporteure nous le rappelait : les avoirs criminels ne sont pas systématiquement identifiés. De plus, environ 30 % seulement des biens saisis finissent par être effectivement confisqués par une juridiction de jugement. Néanmoins, en France, la saisie d’avoirs criminels est en forte progression : en 2011, 109 millions d’euros étaient saisis, contre 771 millions d’euros – dont 27 millions à Marseille – dix ans plus tard, en 2022, soit sept fois plus.

L’argent bien mal acquis […] va enrichir l’État. C’est un juste retour des choses. » À Marseille, il y a un an, une maison ayant appartenu à des narcotrafiquants définitivement condamnés a fait partie des premiers biens immobiliers saisis par la justice en France et a été confiée à une œuvre sociale.

La contestation des décisions de saisie représente actuellement 40 % du contentieux dans certaines chambres de l’instruction. L’article 1 permet ainsi d’alléger le contentieux tout en autorisant les contestations auprès du premier président de la cour d’appel. Dans cette même veine, nous accueillons favorablement les précisions apportées en commission à l’article 3 afin de simplifier les procédures qui enrayent parfois la machine sans pour autant obérer les droits du justiciable.

En plus de ces propositions, nous nous associerons aux améliorations, en particulier celles qui concernent les modalités d’attribution des biens confisqués. Chers collègues, ce texte est une avancée qu’il nous plaît de saluer dans cet hémicycle : au delà du tout prison,

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la saisie et la confiscation ont longtemps joué un rôle secondaire au regard des peines principales que sont l’emprisonnement et l’amende. Cette peine accessoire s’est cependant progressivement installée comme instrument répressif en Europe depuis le milieu des années 1980. En Italie d’abord a été votée en 1982 la loi Pio La Torre, du nom du célèbre député communiste sicilien qui paiera de sa vie la lutte contre la mafia et laissera en héritage le premier dispositif de confiscation obligatoire des biens criminels. En France, il faudra attendre 2010 et la loi défendue par le député Jean Luc Warsmann pour que soient mis en place les outils permettant la confiscation des avoirs criminels par les juges, notamment l’Agrasc. Cette nouvelle politique publique de confiscation

Puis, en 2021, deux textes sont venus compléter cet arsenal, en facilitant la saisie et l’affectation sociale des biens immobiliers confisqués et en instituant un mécanisme de restitution des biens mal acquis l’aide au développement. Ainsi, depuis quatorze ans, la confiscation des avoirs criminels s’est développée en France et a permis de frapper les acteurs de la criminalité organisée beaucoup plus durement que par des peines d’emprisonnement. On peut se satisfaire grandement de l’ensemble de ces dispositions et de la première décennie d’existence de l’Agrasc, mais plusieurs axes d’améliorations demeurent. Certaines activités criminelles continuent à rapporter gros. Je pense, par exemple, au trafic d’armes, à la cybercriminalité, à la criminalité environnementale, mais aussi au trafic de drogue. À cet égard, le directeur général de la police nationale indiquait lors de son audition par la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic que celui ci générerait des gains d’environ 3 milliards d’euros annuels dans notre pays. L’essentiel de l’énergie des pouvoirs publics doit être utilisé pour s’attaquer à ce pactole. En effet, ces activités ont des effets désastreux. Les règlements de compte laissent de trop nombreuses familles endeuillées. Des milliers de policiers et de magistrats mobilisés luttent quotidiennement contre ces trafics. Nous devons les accompagner.

condamné d’un réseau criminel a la possibilité de conserver ses biens dès lors que les juges n’ont pu prouver que ceux ci sont le produit de l’infraction. Autant dire que le crime paie encore et que les sanctions existantes ne sont pas assez dissuasives. Si les délinquants représentent parfois un modèle pour des jeunes, c’est aussi parce que leur enrichissement n’est pas assez remis en cause. À cet égard, malgré une progression fulgurante des confiscations, nous demeurons loin des résultats atteints par l’Italie, ce pays ayant confisqué pour plus de 11 milliards d’euros de biens à la mafia au cours des vingt dernières années et généralisé leur usage social. social. En 2019, 947 biens criminels y ont été mis au service de l’économie sociale et solidaire, par l’intermédiaire de 505 associations ou organismes d’HLM, de 26 fondations, de 27 écoles, de 16 associations sportives ou encore de 5 organismes de formation professionnelle.

que les systèmes mafieux ne l’emportent pas sur la défense du bien commun. C’est ainsi que nous réparerons nos territoires des dommages commis par le crime. Enfin, le plein succès de ce nouvel arsenal ne sera atteint que lorsque l’ensemble des acteurs de la justice auront eux mêmes pleinement intégré une peine de confiscation, devenue le pivot de la lutte contre les phénomènes criminels organisés, et qu’ils auront renouvelé leur approche de la sanction pénale en ce domaine. Aujourd’hui, de nombreuses juridictions n’ont pas recours aux pratiques de confiscation, car celles ci sont chronophages et requièrent une certaine technicité. Nous devons donc les accompagner. Vous l’aurez compris : nous sommes de ceux qui croient que ce qui fait l’efficacité de la peine et la rend dissuasive est non pas sa sévérité, mais sa certitude.

Pour y parvenir, il revient notamment au législateur de rendre plus efficace l’application des mécanismes de saisie et de confiscation des avoirs criminels. En 2010, il y a presque quinze ans, la loi Warsmann avait marqué un tournant dans le domaine de la saisie criminelle. Notre pays s’était doté d’un dispositif normatif important en matière de saisie et de confiscation des avoirs criminels, offrant de larges possibilités opérationnelles et permettant de prononcer des sanctions patrimoniales significatives. Comme souvent, lorsque le législateur introduit de nouvelles mesures, il est bon d’y revenir quelques années plus tard afin d’ajuster et de renforcer certaines d’entre elles ou, au contraire, d’abandonner celles qui ne fonctionnent pas.

Je salue leur travail, car le domaine abordé n’est pas à la portée de chacun et il est impératif que nos réflexions et nos prises de position s’élaborent en en ayant une connaissance suffisante.

Ce qui a été institué en 2010 est performant, mais il n’est pas encore un réflexe pour les acteurs judiciaires, qui n’y recourent que dans des domaines trop spécifiques. Les parquets constatent que les saisies sont largement circonscrites à la délinquance et à la criminalité organisées, qui se révèlent, plus que d’autres, génératrices de profits pour leurs auteurs. revanche, dans la délinquance dite de moyenne intensité, il est à déplorer que le dispositif législatif, pourtant largement applicable, demeure trop rarement utilisé.

et la portée de ces différentes dispositions. Nous saluons naturellement l’ensemble des avancées de nature à faciliter l’action des enquêteurs, des magistrats et de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Qu’il s’agisse de rendre systématique la notification à l’Agrasc de toutes les saisies effectuées et de toutes les décisions de confiscation prises par les juridictions de jugement ou encore d’étendre la compétence de cette agence aux biens non restitués, ces mesures vont dans le bon sens et contribueront à renforcer l’efficacité générale du dispositif de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Nous saluons également les dispositions de l’article 3, ainsi que les améliorations apportées par notre rapporteure. Je pense notamment à la confiscation systématique et de plein droit des biens lorsqu’ils « ont servi à commettre l’infraction, ou étaient destinés à la commettre ou sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction Je me réjouis de l’adoption d’un amendement que j’avais déposé en commission et qui tend à prévoir l’affectation des biens immobiliers saisis et confisqués aux services d’enquête, aux services judiciaires, à l’Office français de la biodiversité ou à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Nous ferons de nouveau des propositions par le biais d’autres amendements afin de contribuer à l’amélioration de ce texte. Il n’en demeure pas moins que ces dispositions participent

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la semaine dernière, j’intervenais à cette même tribune dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille. L’objectif de ce texte était de faire en sorte que se vérifie, même en matière matrimoniale, le principe selon lequel le crime ne paie pas. En matière pénale, ce principe revêt une importance d’autant plus capitale qu’il conditionne à la fois la crédibilité et l’efficacité de la réponse pénale. pénale. Selon l’ancien principe de droit romain, nul ne doit tirer profit de son délit. Aussi, les dispositifs de saisie et de confiscation qui permettent d’appréhender les biens issus ou en lien avec des activités délictuelles sont des leviers puissants de lutte contre la délinquance et la criminalité organisée. Il apparaît en effet que les acteurs craignent davantage qu’on s’en prenne à leur portefeuille qu’à leur liberté. C’est tout le sens de la proposition de loi que nous examinons, qui vise précisément à améliorer l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Je salue le travail important de son auteur, le député Jean Luc Warsmann, ainsi que son engagement remarquable sur ce sujet, puisque c’est à lui que l’on doit la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. C’est en effet en grande partie sur ce texte que repose notre système actuel de saisie et de confiscation, notamment la création de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui joue un rôle essentiel en assurant la gestion des biens concernés. Ce système, tout comme la philosophie qu’il sous tend, se révèle d’une efficacité redoutable, puisque le nombre et le montant des saisies et des confiscations réalisées sont en constante augmentation. Ainsi, en 2023, le montant des saisies réalisées dépassait les 1,4 milliard d’euros, soit une augmentation de 87 % par rapport à l’année 2022, tandis que le montant des confiscations atteignait les quelque 175,5 millions d’euros. Si ces résultats sont encourageants, d’importantes marges de progression subsistent. On estime, par exemple, que seuls 30 % des biens saisis finissent par être effectivement confisqués. Aussi faut il se donner les moyens de frapper encore de frapper encore plus fort le patrimoine des délinquants, afin de les priver du fruit de leurs infractions. À cette fin, le texte met en œuvre certaines des recommandations d’ordre législatif formulées par la mission d’évaluation conduite en 2019 par les députés Jean Luc Warsmann et Laurent Saint Martin. Certaines de ces recommandations ont en effet déjà été satisfaites, telles que la possibilité de réaffecter les biens confisqués ou la prise en compte des tiers dans la procédure de confiscation. Concrètement, la proposition de loi que nous examinons s’organise autour de trois axes : l’amélioration du fonctionnement de l’Agrasc, l’élargissement des possibilités d’affectation des biens saisis et confisqués, et l’aménagement de la procédure pénale applicable aux saisies et

Les juges auront désormais l’obligation de confisquer les biens qui sont l’objet, le produit ou l’instrument de l’infraction. Composé initialement de trois articles, le texte a substantiellement été enrichi

qui est la maison des collectivités. La commission des lois de notre assemblée a salué un ensemble de mesures pragmatiques, qui visent essentiellement à faciliter le travail des enquêteurs et à renforcer l’efficacité des mécanismes de saisie et de confiscation, en conformité avec les besoins exprimés

Son travail a permis d’aboutir à certaines modifications visant à faciliter l’appropriation par les acteurs des nouveaux outils créés par le texte. Il en va ainsi des précisions apportées concernant la confiscation obligatoire figurant à l’article 3. Au terme de son examen en commission, celle ci emporte désormais l’absence d’obligation de motivation, ce qui est cohérent avec l’objectif poursuivi de plus grande efficacité du dispositif. En outre, alors que ce même article précise que la confiscation titre d’expulsion, un amendement adopté à l’Assemblée nationale a étendu la portée de cette expulsion, non seulement à la personne condamnée, mais aussi à tout occupant de son chef. La rapporteure a apporté à ce dispositif une précision de bon sens, en prévoyant que la procédure d’expulsion, prévue à l’article 3, ne puisse pas viser des locataires légitimes, de bonne foi, étrangers aux agissements du condamné. En visant à permettre aux mécanismes de saisie et de confiscation des avoirs criminels, véritables instruments de politique publique, d’atteindre leur plein potentiel, ce texte témoigne d’une forte volonté de renforcer l’efficacité de notre justice et sa réponse pénale.

L’un d’entre eux me permet d’aborder la proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels qui nous est aujourd’hui soumise. Plusieurs témoignages sont allés en effet dans le même sens : la prison ne constitue plus une menace suffisante pour bon nombre de criminels liés au narcotrafic. « Le seul moment où on les voit pleurer, c’est quand on saisit leur appartement, leur compte en banque ou leur voiture Cette phrase revient souvent chez les policiers, les gendarmes, les douaniers ou les magistrats rencontrés. D’ailleurs, plusieurs médias ont rendu compte, après l’opération « place nette XXL » menée à Marseille, de commentaires bravaches de dealers depuis leur cellule. Ces épisodes ont marqué l’opinion : les dealers continuaient de se moquer de la société et de gérer leurs affaires depuis la prison. Rassurons les, il existe des moyens de leur faire mal. Il s’agit de les frapper au portefeuille, car si la détention est parfois perçue comme une période de formation continue durant laquelle les affaires continuent de prospérer, les saisies et confiscations représentent une véritable remise en cause de la pyramide des valeurs sur lequel repose le monde des narcos. En vérité, cette indifférence supposée à l’égard de la détention – car je veux croire qu’il y a aussi une part de mise en scène dans cette fierté déplacée – n’est pas le fait du seul monde des narcos. J’en veux pour preuve plusieurs scènes d’une série inspirée par une enquête de Fabrice Arfi,, de Fabrice Arfi,, qui évoque l’arnaque du siècle, la fraude à la TVA sur les quotas de carbone. Pour ne pas divulgâcher l’essentiel de l’intrigue, je me contenterai de dire que les personnages de ce psychodrame semblent n’avoir pas beaucoup de craintes quant au fait d’être incarcérés : ce qui les inquiète au premier chef, c’est de perdre le fruit de leur illégal labeur. C’est tout l’enjeu du texte examiné aujourd’hui : il s’agit d’éviter que « le crime paie », pour reprendre un titre célèbre du rap français. En la matière, notre pays ne part pas de rien. l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a revendiqué un montant de saisies réalisées en hausse, dépassant 1,4 milliard d’euros, ce qui représente une augmentation de 87 % par rapport à l’année précédente. Le montant des confiscations a également augmenté, pour atteindre 175,5 millions d’euros

prévoit quelques mesures techniques qui permettront sans aucun doute de lever certaines réticences ou craintes chez les magistrats. Mais le nerf de la guerre se situe aussi ailleurs : en ce qui concerne les axes d’amélioration des saisies, un consensus a émergé pendant les auditions de la rapporteure Muriel Jourda sur la nécessité d’une meilleure identification des

parce qu’il nous semble normal d’entendre aussi les propositions de la société civile en matière de lutte contre le crime organisé. À cet égard, je signale notre amendement visant à rendre obligatoire la confiscation de biens en cas de délit ou de crime puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Issue de l’Assemblée nationale, cette proposition de loi s’ajoute à la liste des nombreuses initiatives menées sur ce sujet par les députés Warsmann et Saint Martin, dont nous tenons à saluer la rigueur et la précision du travail. travail. Mes chers collègues, il est tout bonnement insupportable de constater que seuls 30 % des biens saisis finissent par être effectivement confisqués par une juridiction de jugement, à cause de difficultés persistantes à identifier, de manière systématique, les avoirs criminels. Je rappelle que le chiffre d’affaires annuel du trafic de drogues en France est estimé à 3 milliards d’euros. Si la grande majorité des dispositions de ce texte peuvent apparaître, de prime abord, comme de nature essentiellement technique, répondent en réalité à des impératifs simples et indispensables. Le produit du crime doit profiter à la collectivité et être mis au service de l’intérêt général. L’examen de ce texte est l’occasion de rendre hommage à l’action quotidienne et déterminée des enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales, des services des douanes, des magistrats, et bien sûr de l’Agrasc. Pour l’année 2023, le montant des saisies réalisées dépasse 1,4 milliard d’euros ! Cette somme, loin d’être négligeable, est d’une importance majeure, au regard de l’état particulièrement dégradé de nos finances publiques…

Par ailleurs, nous souscrivons pleinement à la modification apportée par la commission à l’article 1 C visant à recentrer la notification à l’Agrasc des décisions de saisie et de confiscation sur celles qui entrent dans le périmètre de ses compétences. Nous éviterions ainsi que cette agence se trouve noyée sous une masse de décisions qu’elle ne pourra ni exploiter ni conserver et qui n’auront pas d’intérêt opérationnel. Il en est de même de l’extension aux CJIP en matière environnementale de la possibilité, prévue dans le texte pour les CJIP classiques, d’obliger la personne morale mise en cause à se défaire de tout ou partie des biens saisis pendant la procédure. Sur proposition de la rapporteure, nous permettrons également aux officiers de police judiciaire de procéder, sur autorisation d’un magistrat, à certaines saisies spéciales nouvelles. Notre lutte contre la délinquance, et singulièrement contre la criminalité organisée, ne doit pas faiblir. Il faut frapper au portefeuille les délinquants, pour qui les gains rapides et faciles sont encore trop attractifs. Aussi, le groupe Les Républicains est pleinement satisfait des modifications apportées au texte par notre rapporteure, Muriel Jourda, dont je salue la qualité du travail mené sur un sujet essentiel,

5 millions de consommateurs réguliers de cannabis et 600 000 usagers de cocaïne, les stupéfiants rapportent environ 3 milliards d’euros chaque année aux trafiquants. Dans ces conditions, la ponction financière est la meilleure des sanctions

permet la mise à disposition des biens immobiliers saisis ou confisqués au secteur associatif ou à des organismes concourant à la politique du logement, à la suite du rapport de Laurent Saint Martin et Jean Luc Warsmann, seuls 30 % des biens concernés sont finalement confisqués. Nous devons aller plus loin, beaucoup plus loin. Quels sont les apports de la présente proposition de loi ? Le texte que nous examinons vise à mieux identifier ces avoirs pour mieux les saisir. pour mieux les saisir. Les gendarmes et les policiers pourront réaliser des enquêtes patrimoniales destinées à priver les malfaiteurs de tout profit. La présente proposition vise également à améliorer l’emploi de ces avoirs criminels. Elle permet à de nouveaux organismes d’en bénéficier, notamment à l’Agence française pour la biodiversité, grâce à un amendement de nos collègues Nathalie Delattre et Paul Toussaint Parigi. et Territoires est particulièrement favorable à la possibilité offerte aux collectivités territoriales de bénéficier de la mise à disposition gratuite des immeubles saisis ou confisqués. Une autre disposition du texte simplifie les procédures d’expulsion des immeubles faisant l’objet d’une décision de confiscation. La confiscation, et c’est très important, vaudra désormais titre d’expulsion de la personne contre laquelle elle est rendue et contre tous les occupants de son chef. Cette solution permettra d’accélérer les procédures ainsi que la mise à disposition de ces immeubles confisqués au profit des victimes ou de l’intérêt général. Le texte corrige également certaines anomalies. Le droit actuel ne permet la restitution des biens mal acquis que lorsqu’ils font préalablement l’objet d’une cession. Cela empêchait précisément la restitution de sommes d’argent saisies. De même, les biens saisis ne donnent pas tous lieu à confiscation, certains d’entre eux étant restitués, d’autres restant dans les limbes, saisis, mais non confisqués ni restitués. Il était important de donner une affectation à cette catégorie de biens : la proposition de loi prévoit qu’ils pourront désormais être employés pour indemniser les victimes.

Elle a notamment introduit la possibilité pour les officiers de police judiciaire de saisir plus rapidement les biens afin qu’ils ne disparaissent pas. La confiscation pas. La confiscation des avoirs criminels pose des questions d’efficacité et de justice. Il n’est pas facile de mettre en œuvre un mécanisme parfait de confiscation des biens.

effet, la question de la confiscation se pose de façon prégnante à cause des avoirs russes gelés. Ce texte pourrait être le moyen d’imprimer la culture juridique française aux textes européens en préparation.

pour qu’un châtiment produise l’effet voulu, il suffit qu’il dépasse l’avantage résultant du délit ». Comme le rappelait Beccaria, l’efficacité d’une sanction tient en grande partie à son caractère dissuasif. Les délinquants, bien plus encore que de leur liberté, à tout le moins autant, redoutent surtout d’être privés du fruit de leurs crimes. C’est sur le fondement de cette philosophie et fort de l’exemple italien qu’une étape symbolique a été franchie en 2010 avec l’adoption de la loi Warsmann, qui a sanctuarisé la culture de la confiscation des avoirs criminels. Alors que les peines privatives de liberté ne constituaient plus, à elles seules, une réponse suffisamment efficace à la lutte contre les réseaux de trafiquants, elle a veillé à armer la justice d’un cadre procédural spécifique. La culture de la confiscation des avoirs criminels en France s’est exprimée dans cette loi. Elle a permis d’élargir le champ des biens susceptibles d’être saisis et confisqués, de clarifier les procédures pénales applicables et d’améliorer la gestion desdits biens, notamment par la création de l’Agrasc, l’une des avancées les plus significatives. Depuis la création de ladite agence, et sous l’effet du renforcement de l’arsenal juridique mis le nombre et le montant des saisies et confiscations qu’elle a réalisées attestent du succès de cette dynamique vertueuse. Ainsi, alors qu’en 2011 le montant des biens saisis s’est élevé à 109 millions d’euros, il est passé à 1,4 milliard d’euros, en 2023. Les confiscations d’actifs ont, quant à elles, explosé, passant de 700 000 euros en 2011 à 175 millions d’euros en 2023. Si nous pouvons nous féliciter de cette progression notable, nous demeurons loin des résultats atteints par l’Italie, qui a confisqué plus de 11 milliards d’euros de biens à la mafia au cours des vingt dernières années et qui en a généralisé l’usage social.

Au moment où certains magistrats réclament la mise en place d’un plan Marshall contre des réseaux disposant de moyens financiers, technologiques et humains considérables, le texte que nous examinons rappelle ô combien ! que la saisie et la confiscation des gains criminels constituent l’un des moyens nécessaires, sinon essentiels, pour priver la criminalité organisée des ressources qui lui permettent de prospérer.

L’évolution de la grande criminalité organisée et internationale doit indéniablement conduire le législateur à mettre en place des dispositifs pour la combattre, sinon à armes égales, du moins avec une efficacité suffisante. C’est cette impérieuse nécessité qui nous amène aujourd’hui à compléter le cadre procédural élaboré en 2010, qui tend à donner force de droit à l’adage bien connu : nul ne doit tirer profit de son délit. À cet égard, le texte qui nous est soumis permettra notamment d’améliorer la gestion des biens saisis et de mieux maîtriser les frais de justice. Il vise également à simplifier l’indemnisation des victimes dans la gestion des biens confisqués, ainsi qu’à renforcer l’efficacité des condamnations pénales. Il prévoit de renforcer la formation des magistrats et des personnels des services de police judiciaire.

afin de frapper de manière irréversible l’accumulation des patrimoines et de développer les possibilités de confiscation. La confiscation obligatoire des avoirs criminels en cas de condamnation pénale doit donc être la pierre angulaire de la lutte contre les organisations criminelles et être davantage mise en avant. Aussi ai je proposé avec plusieurs de mes collègues un amendement visant à renforcer cette confiscation en la rendant obligatoire, même lorsque l’origine des biens

ce texte permet des avancées nécessaires et attendues non seulement de la plupart des acteurs de la justice, mais aussi de l’Agrasc en matière de saisie et de confiscation. Tout en préservant les garanties procédurales offertes aux mis en cause, il donnera une plus grande effectivité au principe selon lequel une sanction pénale doit s’accompagner de la privation du bénéfice de l’infraction commise. Pour toutes ces raisons, le groupe Union Centriste votera en faveur de cette proposition de loi. La parole

accordons à dire que la question des saisies et des confiscations est au cœur de la lutte contre la délinquance et contre la criminalité organisée, mon propos portera sur les moyens et les axes d’amélioration de la réforme de la police judiciaire. Le rapport d’information de Nadine Bellurot et Jérôme Durain,

Si un consensus a émergé sur la nécessité d’une meilleure identification des avoirs criminels dans le cadre des saisies, les moyens et les effectifs manquent cruellement,

en matière économique et financière. Les effectifs consacrés au traitement des contentieux économiques et financiers, qui interviennent également sur les enquêtes patrimoniales, sont insuffisants et leur champ d’action est en souffrance au sein de la police judiciaire : Outre un processus administratif parfois trop lourd, il apparaît donc que des équipes dédiées doivent être créées et que c’est en ce sens que la PJ doit être réformée. C’est notamment le cas pour le traitement des contentieux en matière économique et financière, propos desquels l’autorité judiciaire se trouve régulièrement en difficulté pour saisir un service spécialisé. Un rééquilibrage des moyens entre voie publique et investigation est donc indispensable. Cela suppose une augmentation proportionnelle des moyens renforcés aux personnels réalisant des missions de police judiciaire au sein de la police nationale. dite Lopmi, la filière investigation a obtenu des résultats dans l’exercice des missions d’investigation des forces de sécurité intérieure et a aussi renforcé l’efficacité de leur action, tout en offrant de meilleurs services aux citoyens, il est important de rappeler la nécessité d’inscrire la filière investigation dans le long terme, en construisant de véritables parcours de carrière avec la nécessaire évolution des services d’investigation numérique, notamment de nouveaux outils technologiques.